Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, le budget de la mission « Action extérieure de l'État » est au coeur des missions régaliennes de l'État puisqu'il finance l'action diplomatique de la France, mais aussi sa politique d'influence culturelle et les services consulaires aux Français de l'étranger. Contrairement aux autres missions régaliennes, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une légère baisse des moyens dédiés à la mission « Action extérieure de l'État » en 2018. Les crédits prévus s'élèvent à 3 milliards d'euros, ce qui correspond à une diminution d'environ 0,1 % en valeur et de 1 % en volume en tenant compte de l'inflation. L'exercice 2018 sera donc marqué par la poursuite des efforts budgétaires réalisés ces dernières années. Dans l'ensemble, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères fait preuve de sérieux budgétaire- il faut le noter -et contribue à l'effort de redressement des comptes publics. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit également une diminution des crédits de 110 millions d'euros en 2019- vous semblez étonné, monsieur le ministre, mais je ne fais que rappeler la loi de programmation, qui a prévu des efforts importants sur ce budget ! -et de 65 millions d'euros en 2020, ce qui correspond à une baisse cumulée de 6 % entre 2018 et 2020. Cette trajectoire de dépenses suscite de véritables interrogations compte tenu des engagements du Président de la République à pérenniser certains budgets, par exemple en faveur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, ou des bourses d'enseignement supérieur.

Pour revenir au projet de budget pour 2018, mon examen a porté plus spécifiquement sur le programme 105, qui concerne les dépenses de personnel et de fonctionnement du réseau diplomatique et les contributions internationales, et le nouveau programme dédié à la préparation de la présidence française du G7.

une baisse des contributions internationales de 11 millions d'euros et la stabilisation des contributions aux opérations de maintien de la paix. Il faut enfin relever la poursuite de l'effort budgétaire en matière de lutte antiterroriste et de sécurisation des implantations du ministère à l'étranger

En revanche, plusieurs sujets appellent à la vigilance et mériteront des travaux plus approfondis de la commission des finances dans les mois à venir. Tout d'abord, malgré les mesures entreprises pour adapter le réseau aux priorités diplomatiques de notre pays, certains postes demeurent mal dimensionnés Le processus de mutualisation et de colocalisation, que ce soit avec l'Allemagne, mais aussi avec les délégations de l'Union européenne, doit être poursuivi, voire, si c'est possible, accéléré et amplifié. Des synergies avec les autres administrations de l'État présentes à l'étranger peuvent aussi être trouvées. Ensuite, la politique immobilière du ministère se trouve dans l'impasse sous l'effet de l'érosion des produits de cession. Avec un patrimoine immobilier estimé à 4,3 milliards d'euros à l'étranger et à environ 500 millions d'euros en France, les dépenses d'entretien sont croissantes. Or, parallèlement, les produits de cession diminuent- seulement 30 millions d'euros attendus en 2017. Un rattrapage est espéré en 2018, mais de grandes incertitudes subsistent, comme toujours en matière de cession. Enfin, le mécanisme actuel de couverture du risque de change est incomplet. Les ordres d'achats à terme effectués par l'Agence France Trésor pour le compte du ministère devraient permettre d'enregistrer un gain d'environ 30 millions d'euros en 2018.

Un rapport d'inspection sur le risque de change a été remis au Parlement il y a plus d'un an. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous en dire plus sur l'avancée des travaux et sur les objectifs de votre ministère en la matière ?

Une enveloppe globale de 36 millions d'euros est prévue pour 2018 et 2019. Cette estimation se fonde sur le coût du G20 de Cannes de 2011, en tenant compte des frais supplémentaires liés aux réunions ministérielles et de l'inflation. Le choix du site du sommet déterminera en grande partie son coût final. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement d'appel sur ce point. Dans l'ensemble, le budget proposé pour 2018 donne des gages de sérieux et apparaît équilibré. Un geste ponctuel en faveur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger serait sans doute nécessaire ; c'est pourquoi Rémi Féraud et moi-même vous présenterons un amendement en ce sens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues, à la suite de Vincent Delahaye, je vais vous présenter les programmes de la mission « Action extérieure de l'État », qui concernent les Français à l'étranger et les affaires consulaires, d'une part, la diplomatie culturelle et d'influence, d'autre part. Ceux-ci représentent environ un tiers des crédits de la mission. Le premier constat à la lecture du projet du Gouvernement est la globale stabilité de la prévision budgétaire pour 2018 par rapport à l'année 2017, comme l'a souligné mon collègue Vincent Delahaye. Elle devrait permettre de couvrir les besoins de l'administration consulaire, du réseau culturel à l'étranger et des opérateurs. Mais si ce budget ne présente aucun sacrifice sur les missions essentielles de service public et de diffusion de la culture, et de la langue françaises- hormis l'enseignement français à l'étranger, j'aurai l'occasion d'y revenir -, aucune ambition véritablement nouvelle n'est affichée non plus. Or la situation financière des acteurs culturels et des opérateurs chargés de la politique d'influence de notre pays demeure fragile. Il sera donc, au-delà de cette année 2018, nécessaire d'établir une stratégie claire de développement du français. Le Président de la République, dans son discours du 2 octobre dernier devant l'Assemblée des Français de l'étranger, a fait un certain nombre d'annonces qui semblent aller dans ce sens. Néanmoins, elles ne se traduisent pas par un effort particulier inscrit au budget de 2018. Nous ne pourrons donc juger de l'action du Gouvernement dans ce domaine qu'à l'aune du budget 2019 et des suivants du quinquennat. Certes, la volonté affichée ces cinq dernières années de promouvoir l'attractivité touristique de la France est confirmée : la reconduction des moyens de l'opérateur Atout France est une bonne nouvelle, tout comme la stabilisation des crédits alloués à l'Institut français, aux instituts français et aux alliances françaises. Cependant, ces derniers restent dans l'attente de la mise en oeuvre d'une nouvelle impulsion en faveur de l'influence culturelle et de la promotion de la langue française. Là encore, un plan doit être annoncé au premier semestre 2018, à la fois pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme dans le monde, ainsi que sur un possible rapprochement entre l'Institut français et la Fondation Alliance française. L'exercice 2018 sera également marqué par la poursuite des chantiers de modernisation de l'administration consulaire engagés par les gouvernements précédents. La simplification des démarches- demande en ligne des passeports, répertoire électoral unique, vote électronique -doit ainsi permettre de contenir ces dépenses à un niveau équivalent à celui de 2017. Ces signaux positifs sont à saluer, mais ils ne doivent pas pour autant nous faire perdre de vue l'inquiétude des opérateurs, en manque de visibilité par rapport aux années qui viennent. À cet égard, les contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels qui lient l'État et les opérateurs apparaissent surtout comme des contrats d'objectifs sans garantie sur les moyens accordés. Je veux revenir, d'abord, sur la situation de plus en plus préoccupante de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Il s'agit d'un des plus grands réseaux d'enseignement public à l'étranger au monde, ce qui en fait un atout très précieux pour le rayonnement de notre pays. Alors que la Cour des comptes avait déjà pointé sa situation financière précaire dans une enquête remise au Sénat en octobre 2016, l'AEFE a subi une annulation de 33 millions d'euros par le décret d'avance du 20 juillet dernier. Pour y faire face, l'Agence a prévu de relever de 6 % à 9 % la contribution versée par les établissements, ce qui entraînera inévitablement une hausse des frais de scolarité. Par ailleurs, l'Agence a prévu de réduire le nombre de postes d'enseignants d'encadrement qu'elle finance : 80 postes d'expatriés et 100 postes d'enseignants résidents dès 2018 ; 160 autres postes pourraient disparaître aussi en 2019. Or ces suppressions de postes d'enseignants risquent de nuire à la qualité de l'enseignement. De même, la hausse de la contribution des établissements, qui se répercute naturellement sur les familles, sera préjudiciable aux écoles françaises compte tenu du contexte de forte concurrence. Les établissements français à l'étranger étaient d'ailleurs en grève lundi dernier, un mouvement très suivi pour protester contre cette coupe budgétaire, mais aussi pour marquer de véritables inquiétudes quant à l'avenir. Si nous sommes attachés à ce service public exceptionnel de l'enseignement français à l'étranger, cette situation justifie des efforts spécifiques pour en garantir les principes, la qualité et l'attractivité. C'est pourquoi, sur l'initiative de Vincent Delahaye et de moi-même, la commission des finances vous proposera d'adopter un amendement visant à augmenter de 30 millions d'euros la subvention pour charges de service public à l'AEFE afin de compenser, notamment, les effets de la régulation budgétaire intervenue cet été. Je dirai aussi un mot de la situation de Campus France, pour lequel les moyens affichés ne sont pas à la hauteur de nos ambitions en matière d'accueil des étudiants étrangers. Dans le contexte mondialisé que nous connaissons, l'Allemagne, mais aussi de nouveaux acteurs, comme la Chine, la Turquie ou l'Arabie Saoudite, misent beaucoup plus que nous sur leur politique d'influence par leur attractivité auprès des étudiants. Enfin, il faut revenir dans le cadre de ce budget sur les conséquences de la suppression de la réserve parlementaire. Eh oui ! Plusieurs options ont été évoquées pour pallier cette disparition, mais une réserve serait contraire à l'esprit initial de la réforme. Une solution pragmatique, associant les acteurs locaux et les parlementaires et n'entraînant pas de surcoûts administratifs, doit donc être privilégiée. soulève quelques interrogations. Nous nous interrogeons, monsieur le ministre, sur les modalités de sa mise en oeuvre et sur l'implication des parlementaires et des élus consulaires quant à l'attribution de ces crédits. Nous serons évidemment très attentifs à vos réponses sur ce point. Pour conclure, je dirais que ce budget est d'abord un budget de transition. La stabilité constatée des subventions accordées aux opérateurs chargés de mettre en oeuvre la politique d'influence de la France se réalise en effet à un niveau que chacun reconnaît comme insuffisant, et elle ne prend pas en compte les coupes budgétaires décidées cet été. Par conséquent, si la commission des finances a approuvé le budget de la mission, celui-ci devra cependant être suivi d'une vraie stratégie de développement du français. Si nous faisons ce choix, il s'agira alors d'un investissement qui devra s'inscrire dans le budget de la Nation. La parole

Le premier va vous plaire. Le programme 105, que je suis supposé vous présenter, n'est que de 1,9 milliard

la commission de la défense et des affaires étrangères l'a voté à une assez large majorité. Le deuxième message, monsieur le ministre, concerne nos dépenses en devises étrangères. dépenses importantes, notamment, pour couvrir nos contributions obligatoires aux différentes organisations internationales : ONU, OTAN, OMS, UNESCO, etc. Un grand nombre de ces dépenses se font en euros, mais plus encore en dollars.

La sécurité se décline en plusieurs piliers. Le plan de renforcement de la sécurité de nos communautés et intérêts à l'étranger et de lutte contre le terrorisme et la radicalisation bénéficiera de 52 millions d'euros, portant l'ensemble des dépenses de sécurisation à 78 millions d'euros en 2018. S'ajoutent à cela 1,63 million d'euros supplémentaires affectés au Centre de crise et de soutien et 37,23 millions d'euros dédiés à la sécurisation de nos emprises à l'étranger : ambassades, consulats, instituts français, établissements d'enseignement à Cet effort était nécessaire et urgent. Sans doute sera-t-il de long terme. Concernant la coopération de sécurité et de défense, notre « premier bouclier au loin », elle bénéficiera de 2 millions d'euros supplémentaires. Cette coopération interministérielle est spécifique, car elle est pilotée par un comité d'orientation stratégique qui peut infléchir en cours d'année, ce qui est rare, lorsque la situation internationale l'exige, les priorités géographiques et thématiques de cette politique. Elle fait preuve de la réactivité attendue, comme en témoigne la liste de ses priorités pour la fin 2017 et 2018, qui comprend : l'appui à la force conjointe du G5 Sahel, qui s'est vu dotée d'un poste de commandement l'anticipation de la sortie de crise au Levant avec le Liban comme point focal- en 2018, 1,22 million d'euros devraient être consacrés aux actions en faveur

le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'interviens comme rapporteur pour avis du programme 151, qui finance les dépenses du réseau consulaire. Mon propos portera sur les aspects budgétaires. Si la baisse de 4,87 % des crédits de ce programme en 2018 est en grande partie liée à la suppression de l'enveloppe prévue en 2017 pour la préparation des élections, elle recouvre aussi, dans une moindre mesure, une diminution de ses dépenses de personnel des moyens alloués au réseau consulaire. Celui-ci recevra 258,4 millions d'euros en 2018, une enveloppe modeste au regard de l'étendue de son implantation, de la densité de son activité et de la palette des services rendus. L'administration consulaire a fourni beaucoup d'efforts ces dernières années pour se réformer, moderniser ses procédures et dégager des gains de productivité. Elle continue d'ailleurs à le faire, avec le souci constant d'améliorer le service rendu aux usagers. Il lui serait pourtant difficile désormais de faire plus avec moins. La stabilisation des crédits de ce programme est donc une nécessité. Dans le détail, certaines petites augmentations sont consenties en 2018, par exemple au profit des téléprocédures. À l'inverse, les crédits d'intervention pour l'aide sociale sont en légère baisse. Si les montants en jeu sont faibles, il faut rappeler leur importance pour nos compatriotes à l'étranger se trouvant dans une situation difficile et qui n'ont pas accès aux prestations d'aide sociale délivrées en France. Nous avons noté la reconduction à 110 millions d'euros de l'enveloppe destinée aux bourses scolaires. Cette stabilisation est bienvenue après des années de diminution puisque son montant en loi de finances est passé de 125 millions d'euros en 2015 à 115 millions d'euros en 2016, puis à 110 millions d'euros comme les années précédentes, la dotation budgétaire devrait être complétée par un nouveau prélèvement sur les réserves de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. En écho à un débat qui s'est tenu en commission, pourriez-vous nous assurer, monsieur le ministre, le ministre, que ce prélèvement porte bien sur un reliquat de crédits de bourses scolaires et non sur certaines provisions constituées à partir des droits d'écolage perçus par les établissements Grâce à cette soulte, la réévaluation de la dotation budgétaire paraît pouvoir être différée cette année encore. Mais, il faut le dire, elle pourra difficilement être évitée à moyen terme si l'on veut tenir compte de l'augmentation continue du nombre d'inscriptions dans le réseau de l'AEFE et de la forte progression des frais de scolarité. Pour finir, un mot sur les visas, composante particulièrement dynamique de l'activité consulaire. La baisse constatée en 2016, dont on connaît hélas ! les raisons, est semble-t-il derrière nous. Les demandes repartent à la hausse en 2017, laissant espérer une augmentation des recettes et donc un retour pour le programme 151. Un dispositif de retour dont je veux souligner l'intérêt,

européenne sur la protection consulaire. La France, dont le réseau est particulièrement développé, va devoir offrir ses services de protection aux ressortissants européens dépourvus de représentation dans les pays tiers. nous inquiétons de la charge induite par ce nouveau dispositif, non seulement d'un point de vue financier, mais aussi en matière de surcroît d'activité pour nos postes, dont les moyens humains sont, vous le savez, comptés. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister concerne la nouvelle procédure de demande de cartes d'identité, désormais calquée sur celle applicable aux passeports, depuis leur intégration dans le fichier des titres électroniques sécurisés. Si l'on ne peut que souscrire à l'objectif fixé, qui est de lutter contre la fraude documentaire et les risques d'usurpation d'identité, il faudrait aussi renforcer les dispositifs mobiles de recueil des demandes, afin que les Français résidant loin d'un consulat puissent

Puiser dans les réserves des établissements, c'est ponctionner des familles françaises, mais aussi étrangères, avec le risque qu'elles fassent à l'avenir d'autres choix que celui de notre système d'enseignement si elles n'en sont pas sûres. Or sans

l'Institut français. Ses moyens sont stables ; c'est bien, mais insuffisant, on l'a vu lors du récent débat dans cet hémicycle. Depuis l'échec du rattachement du réseau culturel à l'Institut français, la question de la place et du rôle de cet opérateur n'est pas totalement résolue. rapprochement avec la Fondation Alliance française est souhaitable pour créer une nouvelle dynamique. Mais attention, pas pour gérer la pénurie de ressources ! Les moyens d'intervention du réseau culturel diminuent ; c'est regrettable. Ce réseau doit pouvoir compter sur un soutien public

Il est vrai, reconnaissons-le, que nous profitons de la conjoncture politique internationale, depuis l'élection de Donald Trump et le référendum sur le Brexit. Mais nous bénéficions surtout de notre image, de notre histoire, et d'une présence culturelle forte sur tous les continents.

Une mission de réflexion sur la diplomatie économique a été confiée au directeur général de Business France. Nous souhaitons que ce travail permette d'améliorer l'accès aux dispositifs pour les PME, de rénover les outils financiers de soutien à l'export et d'impliquer davantage les territoires. Le tourisme est une dimension clef de notre diplomatie économique. Il représente 8 % du PIB, 2 millions d'emplois et 40 milliards d'euros de recettes annuelles. La situation du secteur touristique s'améliore en 2017, mais elle reste fragile. Le financement de la promotion du tourisme doit être consolidé ; l'État devra, en tout état de cause, mettre de l'argent sur la table pour attirer des cofinancements et relancer l'investissement. Mais nous avons d'autres idées ; nous pensons notamment que d'autres sources de financement doivent être mobilisées. Une réflexion est nécessaire concernant les plateformes internet. Certaines seraient prêtes à contribuer au financement de la promotion du tourisme, à condition de ne pas être immatriculées en France. Cela pose problème. Par ailleurs, les sociétés d'autoroutes, dont les bénéfices se comptent en milliards d'euros, ne contribuent pas à la politique touristique, alors qu'elles en bénéficient largement. C'est anormal. Concernant l'attractivité de notre enseignement supérieur, la stabilisation des crédits des bourses est tardive. Le nombre d'étudiants boursiers du gouvernement français a baissé de 24 % entre 2010 et 2016. La France a reculé d'une place dans le classement des pays d'accueil ; c'est très dommage. L'Allemagne consacre trois fois plus de ressources que nous à ses bourses étudiantes. Oui, nos moyens sont insuffisants, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Enfin, le Président de la République a lancé en juin dernier une invitation à l'intention des chercheurs étrangers. Mais les difficultés sont loin d'être levées pour les établissements, qui doivent trouver des financements et ouvrir à ces chercheurs des postes très concurrentiels,

Il a été l'occasion, monsieur le ministre, de vous faire part de l'inquiétude partagée sur toutes les travées de cet hémicycle, et relative à la trajectoire budgétaire des crédits que la mission « Action extérieure de l'État » consacre à notre diplomatie d'influence. Les crédits du programme 185 sont ainsi passés de plus de 750 millions d'euros en 2012 à moins de 680 millions d'euros en 2017, soit une baisse de presque 10 % en cinq ans. J'ai parlé à cet égard de « quinquennat meurtrier ». Remarquons néanmoins qu'à l'été 2017, c'est votre gouvernement qui, non content d'annuler déjà tous les crédits mis en réserve, a supprimé 33 millions d'euros supplémentaires à l'AEFE. Pour 2018, vous nous proposez d'arrêter cette descente aux enfers. Comment ne pas y être favorable ? Les crédits se stabilisent pour chacun des opérateurs : Institut français, alliances françaises, AEFE, Campus France. Certains jouissent même d'une onction présidentielle, comme l'AEFE, à laquelle le Président de la République a promis une sanctuarisation de ses moyens. Mais peut-on raisonnablement être favorable à la perspective de maintenir ces crédits à un si faible étiage ? Nous en avons longuement débattu en commission, et la réponse n'a pas été simple. Nous avons cependant souhaité prendre acte des propos que vous avez tenus lors du débat sur l'avenir de l'Institut français,

Puissent ces engagements se concrétiser dans les mois et les années à venir ... C'est dans cette espérance que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis, le 22 novembre dernier, un avis favorable,

La Fondation Alliance française est en très grande difficulté financière et son avenir en est directement menacé. Il semblerait que son budget soit largement amputé par des loyers non versés depuis des mois. Quelle réponse, monsieur le ministre, pouvez-vous apporter à cette situation de crise ? Je rentre d'un Je rentre d'un déplacement dans un pays du Golfe ; je peux vous dire que le rôle du réseau des Alliances françaises est primordial pour développer et renforcer l'influence de la France. Monsieur le ministre, la Fondation Alliance française a besoin d'un geste de l'État. Tout à fait ! Bravo

secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat sur les moyens de notre diplomatie est évidemment essentiel. La France a une grande diplomatie, universelle et indépendante, héritée de son histoire, maintenue par son engagement constant au service de la stabilité et de la paix. Dans un monde dangereux et instable, la voix de la France est essentielle. Daech, Crimée, Corée du Nord, Brexit, orientation nouvelle de l'administration américaine : chacune à leur manière, ces ruptures stratégiques nous ont propulsés dans une ère d'instabilité. Tous les repères de l'ordre international établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale semblent aujourd'hui vaciller. Démonstration de la puissance des des États-continents, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran ; émergence africaine ; montée du terrorisme islamiste radical, qui ravage le Moyen-Orient, déstabilise le Sahel, menace le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest affrontement entre chiites et sunnites ; remise en cause des libertés en Turquie ; retour de la force et du nationalisme en Russie ... Et voilà que notre projet européen lui-même est atteint dans sa dynamique et dans son essence, que notre alliance militaire la plus étroite, l'Alliance atlantique, est questionnée. Dans ce monde « zéro-polaire », la France est un partenaire fiable, prédictible, crédible, solide. Rendons-en hommage à nos diplomates. Notre diplomatie indépendante, universelle, qui parle à tous et et s'ingénie à proposer des solutions politiques aux crises, est à la foi crédible et attendue. Encore faut-il, monsieur le ministre, lui en donner les moyens. Tel est le cadre dans lequel prend place l'examen de ce budget, d'un peu plus de 3 milliards d'euros, traditionnellement très contraint par les dépenses obligatoires. Saluons le fait qu'il est globalement stabilisé. Les différents rapporteurs en ont très bien décrit les enjeux ; je me contenterai donc, en complément de leur travail très approfondi, de relever deux ou trois points d'inquiétude ou de vigilance. L'immobilier, Ladislas Poniatowski a bien décrit les failles d'un modèle qui consiste à vendre nos joyaux pour financer l'entretien du réseau. Quand on vend du patrimoine historique pour pouvoir réparer les chaudières et refaire les peintures,

tout emplacement symbolique, car c'est un enjeu d'image pour notre pays ? Nous ne sommes pas obligés de refaire l'erreur du palais Clam-Gallas de Vienne. La mue du réseau diplomatique est en cours. Je veux saluer l'engagement de nos jeunes diplomates, qui se retrouvent dans les postes dits « de présence diplomatique », avec de très petits moyens, un ambassadeur et un cadre de catégorie B, quelques contrats de droit local, et qui font face à un vrai défi. Évidemment, c'était mieux que de baisser pavillon, mais il nous semble que l'on a atteint, avec 25 postes dans ce format, les limites du modèle. Point noir, les moyens de notre diplomatie culturelle et d'influence. Ils sont insuffisants, alors que leur effet de levier en matière de rayonnement est considérable. C'est un outil d'influence politique, économique et culturel. La situation de l'AEFE nous inquiète grandement. À la suite de Robert del Picchia, nous serons très nous serons très nombreux à l'évoquer ce soir. Attention, monsieur le ministre, le risque d'une remise en cause, à terme, du modèle de l'enseignement français à l'étranger est réel. Elle porterait un coup décisif à notre influence culturelle internationale. Je terminerai en appelant votre attention sur une toute petite enveloppe de crédits néanmoins complètement stratégique : la coopération de sécurité et de défense. Ces crédits ont souvent été la variable d'ajustement. Ils sont passés de 106 millions d'euros à 63 millions d'euros en une dizaine Nous l'avons regretté et dénoncé. Cette politique si intelligente, qui consiste à construire les capacités de nos partenaires dans une action préventive, globale et de long terme, voit enfin ses moyens stabilisés. Merci, monsieur le ministre

pour le rayonnement de la France. Plus que jamais, dans ce monde incertain, la voix de la France doit se faire entendre avec force, car elle est partout, grâce à nos diplomates expérimentés, la voix de la paix. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Et reconnaissons-le, malgré les étonnantes polémiques, le dernier voyage du Président de la République en Afrique est une belle réussite. Nous pouvons tous nous en féliciter. Pour autant, avant de vous tresser, monsieur le ministre, cher Jean-Yves Le Drian, une couronne de laurier pour votre action, laquelle semble s'inscrire dans le droit fil de vos succès en tant que ministre de la défense, même d'un ancien monde, permettez-moi de formuler quelques remarques et de pointer quelques inquiétudes. À l'image de l'ensemble du projet de loi de finances, les crédits alloués au ministère de l'Europe et des affaires étrangères sont guidés par le si cher à Bercy : « Faire mieux, avec moins ». Si cette exigence budgétaire est compréhensible, et même souhaitable en certains domaines, j'ai la conviction profonde que l'action extérieure de l'État ne doit surtout pas- ou surtout plus 3 milliards d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, votre budget, monsieur le ministre, est en très léger recul. Certains me rétorqueront que je chipote, que 115 millions d'euros de baisse, c'est finalement bien peu de chose. D'autant que, dans un contexte international complexe, la lutte contre la menace terroriste et l'engagement français contre les périls restent une priorité. Soit ! Toutefois, dans cet ensemble d'une relative stabilité, l'apparition d'un nouveau programme, consacré à la présidence française du G7 en 2019, oblige à l'ouverture d'une enveloppe de 26 millions d'euros, répartis entre 14 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 12 millions d'euros de crédits de paiement, et ce dès 2018. La mise en place de ce programme 347 dans nos chapitres budgétaires n'affecte pas, en principe, les programmes consacrés à l'« Action de la France en Europe et dans le monde

J'ai parlé de léger recul, nul ne cherchera à le nier. J'entends déjà les commentaires convenus. On nous parlera de « corrections à la marge », de « variables d'adaptation », ou encore de « modeste contribution à l'effort collectif

Les prises de parole volontaristes et les poignées de main fermes du chef de l'État sont bienvenues, rassurantes et nécessaires pour les opinions publiques ; mais sont-elles suffisantes pour assurer la pérennité du rayonnement de notre pays ? À l'heure d'une communication mondialisée, la force des images est indiscutable. Cependant, la continuité et la permanence de nos réseaux consulaires et diplomatiques, la force et le dynamisme de ce que l'on appelle si bien « la diplomatie culturelle et d'influence » de la France, tout comme le soutien et l'accompagnement offerts aux Français établis hors de France, sont des pièces essentielles, qu'il importe de ne pas négliger. indispensables pour relayer, dans les meilleures conditions de proximité et d'écoute, nos valeurs universalistes, incarnées avec justesse aujourd'hui par le discours présidentiel. Reconnaissons que le ministère pilotant l'action extérieure de la France a contribué, en pleine responsabilité, en toute sérénité, aux efforts budgétaires tendant au redressement des comptes publics.

L'action extérieure de l'État a contribué au désendettement de la Nation. Cela dit, monsieur le ministre, contenir et réduire des dépenses de fonctionnement, rares sont ceux qui s'y opposent, à moins de vivre à crédit, et de creuser une dette que les générations futures devraient éponger. Sauf qu'il y a dans votre politique l'écho d'une petite musique laissant à penser qu'internet, les échanges par réseaux sociaux et les téléconférences peuvent se substituer au travail, à l'enseignement, à la présence des femmes et des hommes qui portent l'image et l'amour de la France sur les cinq continents. Malgré ces inquiétudes, somme toute légitimes, et malgré mes critiques, j'ai envie de vous faire confiance, monsieur le ministre. À l'approche des fêtes de fin d'année,

développer deux d'entre eux. Le premier est d'assurer la place de notre pays dans le monde en tant que diffuseur d'idées et de création. Pour cela, ce budget s'appuie sur l'annonce d'un plan ambitieux pour la francophonie. En effet, 274 millions de locuteurs parlent notre langue dans le monde. Malheureusement, les opérateurs de développement de la francophonie ont vu leur financement s'amoindrir ces dernières années, les contraignant à recentrer leur action sur les zones déjà fortement francophones. En parallèle, il est confié aux entreprises privées le soin d'exporter le français dans les autres zones. Encore une fois, le service public est supplanté par le privé. Vous le savez, pour notre groupe, c'est un

et la centaine d'emplois supprimés d'ici à 2019. Les conséquences sont attendues : soit les établissements réduisent leurs missions, soit les frais d'inscription pour les familles augmenteront, excluant ainsi les plus fragiles d'entre elles. fragiles d'entre elles. Il n'est pas toujours possible de faire plus avec moins, mes chers collègues. Par ailleurs, la francophonie s'appuie également sur l'Institut français pour l'exportation de biens culturels. Mais avec un emploi supplémentaire et 100 000 euros d'augmentation de budget, les perspectives sont, là aussi, compromises. Prenons pour exemple le livre. Le programme de soutien à la traduction des oeuvres françaises a fait ses preuves, faisant de Paris le troisième exportateur européen. européen. Au vu des contraintes budgétaires et de la montée en puissance de concurrents, comment assurer la pérennité de ce dispositif ? De même, il est regrettable que Campus France voie stagner sa subvention pour charge de service public. La France, malgré de nombreux éléments avantageux-

Par ailleurs, un tiers du budget social des étudiants étrangers est consacré aux programmes d'excellence comme Eiffel, Excellence-Major ou Quai d'Orsay-Entreprises. Si ces programmes sont nécessaires, on peut cependant contester cette stratégie à long terme orientée vers l'élitisme. Pour maintenir notre influence, il est essentiel de réagir face aux stratégies offensives des pays concurrents dans tous les domaines : la Turquie ou l'Arabie saoudite dans l'enseignement supérieur, la Chine et les États-Unis dans l'aide au développement en Afrique notamment, la Russie dans les espaces médiatiques, ou encore le Qatar dans le sport, l'industrie du luxe. Le budget proposé Le budget proposé n'est pas à la hauteur de ces attentes. Le second objectif de notre action extérieure est d'assurer aux Français vivant à l'étranger des points d'accroche avec la France. Là aussi, il est difficile de se satisfaire d'un budget

pas mention des 160 millions d'euros de crédits gelés cet été, et non compensés, ainsi que des baisses prévues pour 2019 et 2020, à hauteur de 176 millions d'euros. La France, troisième réseau diplomatique du monde, paie aujourd'hui les choix budgétaires faits en fermant des antennes diplomatiques et en supprimant des postes. Les conséquences pour nos concitoyens à l'étranger mais aussi pour les étrangers souhaitant venir dans notre pays sont importantes.

l'actualité internationale, depuis l'élection de Donald Trump jusqu'à la situation au Moyen-Orient, rappelle combien le monde est devenu instable et imprévisible. L'action de la France dans le monde est plus que jamais attendue et nécessaire. Dans un contexte mondial dégradé, dangereux, comme le montre une fois encore l'essai balistique nord-coréen de la semaine dernière, le monde a besoin de plus de démocratie, de diplomatie et de dialogue.

Dotée du troisième réseau diplomatique et consulaire, de l'un des meilleurs corps diplomatiques au monde, de relais d'influence culturels, stratégiques et politiques anciens sur tous les continents, la France a toutes les cartes en main pour demeurer une grande puissance de diplomatie et de paix. Néanmoins, nous devons veiller à ne pas prendre pour acquise cette position unique sur la scène internationale. L'histoire nous montre que lorsque nous cessons d'investir dans notre diplomatie et notre action extérieure, notre connaissance du monde s'amoindrit, notre voix s'affaiblit, nos choix politiques, enfin, sont moins fermes et peuvent parfois manquer de jugement. À ce titre, l'affaiblissement continu du Quai d'Orsay et du réseau, y compris culturel, de la France à l'étranger, et ce depuis plusieurs années, est inquiétant. Il faut cesser de considérer notre action extérieure comme une variable d'ajustement, sous prétexte que l'on ne peut pas mesurer précisément ce qu'elle rapporte. Les gains en matière de sécurité collective ou de mobilisation autour des grands enjeux de l'humanité, pour impondérables qu'ils soient, n'en sont pas moins indispensables à notre pays, à l'Union européenne et au monde dans son ensemble. L'accent porté, depuis quelques années, sur la diplomatie économique et le tourisme est également un atout non négligeable pour notre économie et nos entreprises. Je le dis aujourd'hui avec force : notre diplomatie est un actif précieux pour la France, un atout pour l'avenir, non le coûteux vestige d'une époque de grandeur révolue. Or vous semblez, monsieur le ministre, poursuivre la mise en oeuvre de cette logique de rabotage progressif des crédits dédiés à cette mission, une fois corrigés des mesures de périmètre. Si nous croyons souhaitable la rationalisation du système de primes des agents diplomatiques, si des économies de fonctionnement sont toujours possibles, nous estimons que la démarche d'économies structurelles arrive à son terme, sauf à revoir drastiquement notre stature diplomatique.

Nous avons constaté, avec l'élection du Président de la République, que l'image de la France est toujours positive à l'étranger, que sa culture est connue et appréciée. Néanmoins, d'autres pays déploient des efforts colossaux dans ce domaine la Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, par exemple, investissent massivement dans leur réseau culturel à l'étranger et occupent les espaces que nous délaissons. Notre propre réseau, atomisé et en perte de puissance, gagnerait à être rationalisé pour répondre à ce défi. Il pourrait s'appuyer sur une ambition renouvelée pour la francophonie, ambition que le Président de la République semble, heureusement, avoir endossée. Nous devons aussi nous interroger

traitement des questions globales, au premier rang desquelles la sécurité et le climat, qui passe par un renforcement de notre présence dans les institutions multilatérales et un pilotage au plus haut niveau politique. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et elle tient ce rôle avec dynamisme et esprit d'initiative. le retrait des États-Unis, le blocage persistant de la Russie, l'attentisme parfois coupable de la Chine et le relatif effacement du Royaume-Uni, empêtré dans le Brexit, la France a une responsabilité accrue pour maintenir vivantes et efficaces les instances du multilatéralisme,

Nous devrons oeuvrer à la construction d'une véritable politique extérieure commune sur les grands sujets qui touchent à notre sécurité commune, aux crises dans notre voisinage et aux biens communs de l'humanité.

C'est bien ce qui m'interpelle : nous regardons. Certes, nous condamnons. La France est un membre du Conseil de sécurité, elle est l'un des pays détenteurs de l'arme nucléaire, dès lors il est regrettable que sa voix reste ainsi inaudible. Mes chers collègues, il est des moments diplomatiques où la singularité française est nécessaire à la scène diplomatique, il est des moments où elle manque. Nous savons que les politiques diplomatiques fondées sur l'isolement et/ou le mépris tendent à cristalliser les tensions et renforcent l'autorité de ceux que l'on se plaît à faire passer pour « fous ». La situation est telle qu'il conviendrait de s'interroger, sans préjugés, sur les moyens à mettre en oeuvre pour la faire évoluer en profondeur. Pour ma part, je continue à penser que nous devrions favoriser le choix du dialogue avec Kim Jong-un. De la même façon, il importerait de rappeler à nos alliés Américains l'importance et la valeur, en termes de sécurité, des traités relatifs à la non-prolifération des armes nucléaires, qu'ils aient été contractés avec l'Iran ou la Russie. Russie. Pour conclure sur ce point, nous devrions être lucides : les sanctions économiques et financières n'apportent pas les résultats attendus. Ces considérations sur l'importance du multilatéralisme dans le monde étant rappelées, j'en viens maintenant au sujet qui nous préoccupe tous Monsieur le ministre, avons-nous une raison d'être rassurés, comme vous l'affirmez, par le nouveau dispositif de compensation appelé à remplacer la réserve parlementaire à destination de projets à l'étranger ? Avons-nous également des raisons d'avoir confiance en l'avenir de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE ? Pour ma part, je rappellerai simplement que, par un décret de régulation du 21 juillet dernier, le budget de la mission « Action extérieure de l'État » a été amputé de 163 millions d'euros en autorisations d'engagement,

Pourtant, vous avez déclaré que « la diminution de la subvention a été gérée de manière à être sans effet pour la rentrée scolaire 2017 ». Et après 2017 ? La diminution est tellement sans effet » que les lycées français à l'étranger se sont largement mobilisés, le 27 novembre dernier, contre la baisse de la dotation de l'État à l'AEFE et les suppressions de postes. Elle est tellement « sans effet » que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée des Français de l'étranger, ainsi que les associations UFE et ADFE, plusieurs syndicats, les associations de parents d'élèves à travers le monde, les enseignants des lycées eux-mêmes vous ont alerté sur les conséquences de ce désengagement pour les familles et la qualité de l'enseignement. Alors, soit nous n'avons pas compris vos explications apaisantes, soit il y a un problème. Mais, au-delà, le moment n'est-il pas enfin venu d'ouvrir les yeux ? Sérieusement, monsieur le ministre, depuis combien d'années avons-nous ce débat sur l'AEFE, son fonctionnement, ses crédits sans cesse rognés, l'absence d'un véritable rectorat pour garantir la bonne gestion de son corps enseignant ? N'est-il pas temps d'avoir le courage d'avouer que cela ne fonctionne plus ? rapport de la Cour des comptes, qui déplore n'avoir vu aucune évolution depuis celui de 2013, lequel pointait déjà les dysfonctionnements d'aujourd'hui. Ce qui est en cause, c'est le modèle économique de l'AEFE qui, vingt-sept ans après sa création, est comme un malade en fin de vie. Ne sachant plus où chercher de l'argent, elle en est au point d'en extorquer aux lycées et aux autres établissements scolaires qui, eux, ont constitué des réserves. Il n'y a pas de vision à long terme pour l'enseignement scolaire à l'étranger. Celui-ci doit pouvoir se financer autrement qu'en prélevant toujours de l'argent sur les familles, lesquelles supportent aujourd'hui des coûts de plus en plus élevés. En rognant toujours un peu plus sur la dotation d'État, on fait, certes, quelques économies, mais ce sont les familles qui en paient le prix

L'AEFE ne peut, de mon point de vue, continuer à être à la fois opérateur et régulateur de l'ensemble du réseau. Il est contradictoire de prétendre piloter une mission d'intérêt général, d'une part, et de gérer directement des écoles, d'autre part. Le rapport de 2016 de la Cour des comptes relevait que l'AEFE se trouvait confrontée à une concurrence de plus en plus intense sur le marché mondial de l'éducation et à un désengagement financier de l'État, alors que la demande des familles françaises et étrangères s'accroît. La décrue programmée des crédits publics ne pourra pas, à terme, rester sans effets. Notre ambition doit être de créer un nouvel élan en faisant évoluer la structure de pilotage de l'enseignement français à l'étranger. J'appelle donc à une vraie remise à plat au bénéfice des familles et de l'enseignement français à l'étranger. Il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière

de budget de la mission « Action extérieure de l'État » est, selon nous, à la fois réaliste et ambitieux. Il est réaliste, car il prend en considération les nécessaires ajustements budgétaires dans certains secteurs. ambitieux, puisqu'il prévoit une hausse globale des crédits alloués à la mission par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Comme nous pouvons le constater, ce projet de budget maintient l'effort financier engagé l'an dernier en faveur de la protection de nos communautés et de nos intérêts à l'étranger, que de la consolidation des moyens de lutte antiterroriste. Ainsi sera intelligemment maintenu, en 2018, le plan dédié à cet effet, avec une enveloppe de crédits supplémentaires de 52 millions d'euros et 67 équivalents temps plein affectés à la sécurité. Concernant la protection des communautés françaises à l'étranger, il apparaît fondamental de rappeler que l'augmentation des budgets alloués à la sécurisation de nos emprises, en particulier les dépenses de gardiennage et de travaux, est pérennisée 22,16 millions d'euros pour la sécurité des ambassades, consulats et instituts français ; 14,7 millions d'euros pour les établissements d'enseignement à l'étranger ; 1 million d'euros pour les Alliances françaises. qui concerne la protection des communautés françaises à l'étranger, est maintenue l'augmentation des enveloppes pour les biens de première nécessité et médicaments ainsi que les dépenses de crise, notamment celles de fonctionnement de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, la CIAV, tout comme les subventions aux associations aidant les victimes. Nous ne pouvons que nous en réjouir Enfin, s'agissant de la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, le renforcement des crédits d'intervention de la Direction de la coopération de sécurité et de défense, la DCSD, se poursuivra en 2018 : 2 millions d'euros viennent compléter les 9,5 millions d'euros d'augmentation de 2017, postes de coopérant créés en 2017 sont pérennisés, afin de renforcer nos capacités d'appui en Afrique et au Moyen-Orient dans le cadre du plan d'action gouvernemental contre la radicalisation et le terrorisme, Autre point important, la stabilité de la ligne des contributions aux budgets des opérations de maintien de la paix en 2018 est le résultat d'une négociation difficile et d'un important effort de rationalisation réalisé durant le mois de juin afin de réduire la proposition budgétaire initiale du secrétariat de l'ONU. Les contributions européennes connaissent, quant à elles, une légère augmentation par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, du fait d'une hausse du budget du Conseil de l'Europe résultant de plusieurs accords partiels. outre, un programme dédié a été créé pour l'organisation du prochain sommet du G7, présidé par la France, qui se tiendra en 2019. Une enveloppe de 36 millions d'euros est prévue à cet effet. Dès 2018, un certain nombre de dépenses devront être réalisées afin de préparer cet événement : réunions des « sherpas » et autres groupes de travail, premières dépenses de location du futur site et aménagements, tenue de réunions des ministres des affaires étrangères et des finances, frais de fonctionnement du secrétariat général et dépenses de communication. Par ailleurs, l'enveloppe de crédits du protocole augmente de 2,4 millions d'euros, pour couvrir les frais induits par la tenue des sommets de la francophonie en Arménie et France-Océanie à Papeete.

Enfin, nous prenons acte de la mise en place d'une enveloppe de 110 millions d'euros destinée à financer les bourses scolaires pour 2018. La prévision des besoins en matière de bourses scolaires est fondée sur une croissance des frais de scolarité qui a davantage été maîtrisée au cours des deux dernières années.

Vous l'aurez compris, ce budget stabilisé, en légère hausse, est bienvenu. Il marque la volonté du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de mener à bien l'action de notre pays en dehors de ses frontières.

Aussi voudrais-je commencer par saluer vos services, monsieur le ministre, en premier lieu nos ambassadeurs et tous les personnels qui servent au sein des postes diplomatiques. J'ai également une pensée particulière pour nos consuls honoraires. Tous ceux que j'ai rencontrés ont toujours été au rendez-vous pour me permettre d'assurer ma mission dans les meilleures conditions. Je ne voudrais pas que l'on dise que je me permets de les juger en vous confiant que je les trouve souvent excellents. C'est en tout cas ce que je pense, et je ne pouvais commencer mon intervention sans leur exprimer ma gratitude. Je veux également remercier les élus consulaires qui oeuvrent au quotidien sur le terrain au service de nos compatriotes, souvent sans compter leur temps. La France est assurément le pays le plus avancé au monde en matière de représentation démocratique de ses ressortissants établis hors de ses frontières. Souvent, les parlementaires étrangers m'interrogent avec envie, en vue de trouver dans notre système une source d'inspiration. Ils m'offrent ainsi une raison supplémentaire d'être fier de mon pays. de budget global du ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'établit pour 2018 à 4,7 milliards d'euros, dont 3 milliards d'euros seront consacrés à l'action extérieure. La dotation de la mission s'inscrit donc dans la parfaite continuité de la dernière loi de finances du précédent quinquennat.

Sur ce dernier point, il convient de souligner l'effort budgétaire spécifique de 12 millions d'euros prévu en 2018 au bénéfice de l'entretien lourd et courant du patrimoine immobilier du ministère en France et à l'étranger. Compte tenu de l'érosion des produits de cession immobilière, les rapporteurs spéciaux ont attiré notre attention sur l'« impasse » dans laquelle se trouve malgré tout la politique immobilière du Quai d'Orsay. Quelle est, monsieur le ministre, la stratégie à moyen terme du Gouvernement en la matière ? Avant de parler du budget du programme 185, je veux évoquer son action 2, et en particulier l'indicateur 2.1 Appui au commerce extérieur. La visite du président Macron en Afrique nous rappelle que, en 1960, la France représentait 20 % des importations africaines, contre 10 % en 2000 et moins de 5 % aujourd'hui.

Avant de faire leurs valises, vos prédécesseurs nous promettaient 20 milliards d'euros de déficit pour cette année. Ce sera plutôt 44,4 milliards d'euros, plus du double de ce qui était prévu il y a un an. Pour 2018, vous prévoyez 48 milliards d'euros de déficit. Pour 2020, c'est le « pompon » : vos prévisions de solde affichent « non déterminé ». Monsieur le ministre, comment pensez-vous qu'une entreprise privée serait jugée sur les marchés si elle s'avouait incapable de proposer des prévisions à trois ans ? maintenant des programmes 151 et 185 afférents aux réseaux consulaire et culturel. Les crédits du programme 151 sont en effet stabilisés, à hauteur de 368,4 millions d'euros. 185 s'établissent à 717,5 millions d'euros, en légère hausse de 0,3 %. Si l'on fusionnait les deux programmes en un seul pour faire des économies d'échelle, on aboutirait à un programme de 1,085 milliard d'euros.

autant que les budgets cumulés de tout le réseau consulaire, de toute l'action en matière de coopération culturelle, Instituts français et Alliances françaises compris, de l'action audiovisuelle extérieure, du partenariat universitaire et de la diplomatie économique, comprenant l'action touristique d'Atout France. L'enseignement français à l'étranger pèse autant que tout le reste ! Cela coûte moins qu'un Airbus A180 ! J'espère que chacun en prend conscience ... Voilà plus d'un an déjà, la Cour des comptes dénonçait un réseau d'enseignement « fragilisé », et invitait les autorités publiques à « insuffler une nouvelle dynamique Le réseau de l'AEFE plafonne à 495 établissements scolaires et à 342 000 élèves, dont 60 % d'étrangers. On se flatte de le voir progresser de 2 % par an. On claironne que nous sommes le seul pays à bénéficier d'un réseau d'écoles à l'étranger, que nous rayonnons

Pendant ce temps, des dizaines de milliers d'enfants français nés à l'étranger n'ont pas accès à l'apprentissage de notre langue et ne la parlent pas. La compétition est aujourd'hui mondiale, et les marges de manoeuvre de plus en plus contraintes. Notre influence dépendra donc de notre capacité à nous renouveler et à nous mesurer à des pays concurrents de plus en plus innovants, de plus en plus audacieux. Atrophié, le réseau AEFE est condamné àdisparaître. Anticipons donc, monsieur le ministre.Sortons des modes de pensée routiniers et entronsde plain-pied dans l'enseignement libre du XXIsiècle ! Dans un contexte concurrentiel marqué par l'expansion des écoles libres, le maintien de 74 établissements « en gestion directe » n'est plus tenable. Les obstacles administratifs à l'homologation d'une nouvelle école doivent être levés. Je vous propose de revoir votre programme en fixant deux objectifs à notre enseignement à l'étranger viser la maîtrise du français par 100 % des enfants français vivant à l'étranger, en créant un chèque éducation ; doubler le nombre d'écoles françaises d'ici à cinq ans, pour que le réseau compte 1 000 écoles, puis 2 000 écoles d'ici à dix ans, en libérant le système. Créons le nouvel élan que tout le monde attend. J'entends bien les arguments en défense de la « spécificité française » émanant des conservateurs de tous bords, mais maintenir l'universalité de notre diplomatie et les moyens de notre influence est un défi quotidien, sans cesse renouvelé, et la France est aujourd'hui bien mal armée pour le relever, du fait d'un déséquilibre de son budget. À vouloir rayonner avec des chandelles, on en arrive à faire des économies de bouts de chandelles. Nous le verrons au travers des amendements que nous allons examiner.

Lors de son discours aux ambassadeurs, en août dernier, le Président de la République avait cité les trois « D » -défense, développement, diplomatie -comme étant les leviers de la stabilité. Ces propos, qui concernaient l'Afrique, sont valables pour l'ensemble de notre politique étrangère. En effet, notre action extérieure doit être pensée de manière globale. Si les armées nous font gagner les guerres, ce sont la diplomatie et le développement qui nous permettent de conquérir la paix. Dans un monde certes plus durablement pacifié, les défis et les périls ne manquent pas : défi de la sécurité, défi d'une meilleure régulation économique, défi de la démocratie, défi de l'Europe et défi climatique. climatique est assurément le péril auquel nous devons faire face en priorité. Du reste, le précédent gouvernement avait fait de la gouvernance climatique mondiale l'un de ses objectifs prioritaires.

La revue stratégique a montré la diversité des menaces, tant sur le plan géographique que sur celui de la nature des acteurs. Dans un monde interdépendant, la sécurité de notre territoire exige la stabilité internationale. Dans cette perspective, la France mène une politique étrangère active en faveur de la préservation de la paix et s'appuie sur une tradition d'excellence diplomatique. La force d'une politique étrangère consiste justement à ne pas s'appuyer uniquement sur sa force, mais aussi sur sa capacité d'influence. Ce pouvoir de convaincre est le levier permettant de garantir nos intérêts. Pour porter ce message, il nous faut maintenir l'excellence de notre corps diplomatique, tout en l'adaptant aux dynamiques nouvelles des relations internationales. Le gouvernement précédent avait d'ores et déjà engagé une modernisation en ce sens. Il faut néanmoins renforcer la qualité de notre offre consulaire, développer la réputation culturelle de notre pays et améliorer son attractivité auprès des étudiants. l'effort que doit prolonger ce projet de loi. Notre position est simple ; elle se fonde sur la cohérence entre ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui sera fait. Le budget est l'acte politique fondamental. Il permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs et les moyens qui leur sont consacrés. C'est bien cette adéquation qui fonde la sincérité et l'efficacité de l'action politique.

Cette continuité s'illustre avant tout par la stabilité budgétaire en trompe-l'oeil des programmes 105, 185 et 151. Une politique ne peut être faite que de mots, c'est pourquoi je relèverai plusieurs points de vigilance, des premières contradictions entre les objectifs affichés et les moyens alloués. Nos craintes sont d'ailleurs renforcées par les pratiques de Bercy, tel le gel de 700 millions d'euros de crédits dans le budget de la défense. Je crains que la stabilité budgétaire, que nous louons, ne soit que de façade.

n'est qu'apparente ; en fait, elle masque un effet de périmètre, avec la création du nouveau programme pour la présidence du G7. Les effectifs du ministère diminueront de 115 emplois en 2018. Une forte dynamique de réduction des emplois avait déjà été enclenchée. Toutefois, aujourd'hui, nous nous interrogeons : comment concilier l'objectif d'un rayonnement universel de notre dispositif consulaire avec une baisse constante des effectifs Pour répondre aux défis de la stabilité, notre action extérieure doit aussi s'appuyer sur la politique d'influence, qui concerne des champs divers comme l'enseignement français à l'étranger, la diffusion culturelle, linguistique ou scientifique et la promotion du tourisme, champs qu'il est indispensable de couvrir pour que notre pays exerce son influence. Sur ce point aussi, l'écart entre les objectifs affichés et les moyens alloués est flagrant. Comment maintenir notre capacité d'influence quand les opérateurs qui y concourent sont fragilisés ? Les moyens dévolus à l'action culturelle subissent une contraction de 1,6 %, ceux qui sont consacrés à l'Alliance française vont encore baisser, l'audiovisuel public à l'étranger est fragilisé, au moment où son poids comme vecteur d'influence est illustré par les stratégies agressives de nombreux pays. ailleurs, le sous-financement du réseau des opérateurs à l'étranger se poursuit. En effet, si les crédits de l'Institut français augmentent de façon modeste, ceux du réseau continuent continuent de diminuer. Au total, l'Institut français aura perdu 25 % de ses moyens depuis sa création en 2011, sur fond de rapprochement avec le réseau culturel porté par la Fondation Alliance française, laquelle est également en grande difficulté. Devant tant d'incertitudes, devant le décalage entre les intentions et les moyens, le groupe socialiste et

Cette position vise, paradoxalement, à soutenir, monsieur le ministre, votre détermination à obtenir des clarifications de la part du ministère des finances, qui pourrait se préoccuper bien davantage de ceux, militaires ou diplomates, qui oeuvrent chaque jour pour assurer la sécurité de notre territoire.

mais ceux qui s'attendaient à y trouver une traduction budgétaire de la vision internationale esquissée, non sans talent, au gré des déplacements présidentiels ou devant l'Assemblée des Français de l'étranger en seront pour leurs frais.

À titre d'exemple, les crédits du programme 185 avaient diminué de 9,2 % au cours du quinquennat Hollande. Plutôt que de redresser la barre, le Gouvernement a décidé, durant l'été, une annulation en gestion de 60 millions d'euros, aux effets particulièrement désastreux pour l'AEFE. Sur l'ensemble des crédits de la mission, 160 millions d'euros ont été gelés en juillet. Si l'on tient compte de cela et des évolutions de périmètre, c'est un budget non pas stable mais sensiblement en baisse qui nous est proposé, et les projections pour 2019 et 2020 ne sont guère rassurantes

il manque une feuille de route, une vraie stratégie de développement de notre politique d'influence. Notre réseau ne fonctionne pas en vase clos. C'est par sa capacité à engager et à animer des partenariats culturels, scientifiques ou universitaires avec des acteurs locaux qu'il fait grandir notre influence. Cela nécessite évidemment des crédits. Un grand plan de promotion du français et du plurilinguisme a été annoncé, mais, dans le même temps, les subventions aux Alliances françaises diminuent de 11 %. Certes, ce réseau est autofinancé à 96 %, mais c'est justement ce type de modèle qu'il nous faut encourager : investir dans des structures qui, à partir de 1 euro public, seront capables de lever des fonds privés et de vendre des prestations de grande qualité. Il existe aujourd'hui une véritable inquiétude des opérateurs quant à leur capacité de continuer à se développer à moyen et long termes. À l'heure où la concurrence fait rage, en matière tant d'audiovisuel extérieur que d'éducation internationale, nous ne pouvons nous contenter de laisser vivoter nos réseaux. Il faut insuffler un nouvel élan.

Il s'agit d'abord d'un projet de création d'une fondation pour le rayonnement français à l'étranger. C'est un projet déjà ancien. Je remarque que les engagements ministériels de pallier la suppression de la réserve parlementaire, qui avait abondé l'année dernière les crédits de la mission « Action extérieure de l'État renouvelés encore tout récemment par Jean-Baptiste Lemoyne en réponse à mon intervention lors du débat sur l'Institut français, n'ont pas encore trouvé de traduction budgétaire dans le PLF. J'ai donc cosigné un amendement en ce sens, mais nous ne pouvons plus continuer de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il semblerait plus judicieux de créer une fondation, de manière à permettre à l'État d'y investir une somme minimale destinée à servir d'amorce pour lever d'autres fonds, d'origine privée. Il existe aussi un moyen peu coûteux de renforcer l'enseignement du français et en français à l'étranger, tout en ouvrant des perspectives internationales à des jeunes ou moins jeunes. Le volontariat international en entreprise connaît un succès impressionnant pourquoi ne pas en imaginer une déclinaison dédiée à l'enseignement francophone ? Financée par les structures d'accueil et pilotée par notre réseau culturel, elle ne pèserait pas dans le budget de l'État, augmenterait notre exposition internationale et constituerait une belle opportunité pour des Français qui sont, ne l'oublions pas, nos premiers ambassadeurs. Je conclurai en évoquant la situation de nos compatriotes à l'étranger. Là encore, le budget est marqué par la stagnation pas de traduction des engagements présidentiels en matière de modernisation des services consulaires, blocage du Gouvernement sur la question de la CSG et de la CRDS indûment payées par les expatriés, malgré une condamnation européenne, pas d'évolution non plus sur la reconnaissance de la résidence unique en France. Si je me réjouis de l'annonce de la création d'une mission parlementaire sur ces sujets, il ne faudrait pas que cette annonce soit, encore une fois, prétexte à l'inertie. Monsieur le ministre, je vous fais confiance pour avancer sur ces dossiers.

sont en premier lieu celles d'un réseau unique, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui scolarise actuellement 350 000 élèves français dans 137 pays et emploie 21 400 personnes. Il constitue aussi, aux dires de tous, un pilier de notre rayonnement en assurant l'éducation de nombreux élèves étrangers.

Le désengagement de l'État fait peser un risque de déconventionnement, donc de privatisation, des établissements, dont la contribution passerait de 6 % à 9 %. Le manque de visibilité sur les efforts financiers qui leur seront demandés risque d'inciter les familles à choisir une autre école. Si l'État ne peut pas tout, les familles non plus, et encore moins celles, françaises ou étrangères, qui entendent transmettre notre langue et notre culture à leurs enfants. Cette baisse de la dotation entraînera inéluctablement une forte augmentation des frais de scolarité dans de nombreux établissements, qui devront remplacer les professeurs résidants ou détachés par des recrutés locaux. Mais la presse a déjà relevé l'indifférence de Bercy pour un tel mouvement. Je voudrais ensuite évoquer la situation des recrutés locaux qui ne relèvent pas de la législation française. Le projet de loi de finances pour 2018 ne fait pas mention des 80 postes d'expatrié et des 100 postes de résident qui seront supprimés. Sur trois ans, plus de 500 postes disparaîtront et seront remplacés par des enseignants recrutés localement, qui n'ont malheureusement pas toujours les bonnes qualifications, dont le vivier se tarit au fil des recrutements, et qui sont à la charge des établissements.

qu'ils ne nous rapporteront, en matière d'image, de signal négatif, voire de régression, alors même que le Président de la République a affirmé le « souci majeur pour nos compatriotes de l'étranger d'offrir à leurs enfants un enseignement de qualité qui conserve un lien fort avec la France ». Monsieur le ministre,

de notre politique étrangère, qui doit nous permettre de disposer des moyens de faire entendre la voix de la France dans un monde en proie

La protection de nos emprises à l'étranger vient au premier rang de nos responsabilités, à l'égard tant de nos agents que de nos compatriotes ; c'est donc pour moi un impératif absolu. Elle exigeait une planification et une augmentation des moyens : plus de 75 millions d'euros seront consacrés à la sécurisation des emprises de notre réseau diplomatique et consulaire, ainsi qu'à nos établissements d'enseignement à l'étranger et aux Alliances françaises. Protéger les Français à l'étranger implique également un engagement face aux crises internationales qui affectent nos intérêts, à commencer par la menace terroriste qui pèse sur l'Europe et sur la France. du ministère fait partie intégrante de notre stratégie de sécurité et de contre-terrorisme. En appui à nos efforts diplomatiques et militaires, nous devons notamment aider les pays en crise à faire face aux tensions, à développer leur propre sécurité, à se stabiliser puis à se reconstruire, comme aujourd'hui en Irak et en Syrie. Cela relève aussi de la sécurité et de la protection des Français, et c'est pourquoi les crédits de gestion de sortie de crise augmentent de 14 millions d'euros, pour atteindre plus de 86 millions d'euros en 2018. Cet effort devra se poursuivre ; il est indispensable à la crédibilité de notre action diplomatique. Parallèlement, nous développons des outils de prévention qui soutiennent directement nos actions en matière de sécurité nationale. Je pense au budget consacré à la coopération de sécurité et de défense,

et de la lutte contre le trafic de migrants. Enfin, notre sécurité comme le maintien de notre rang international passent aussi par notre action en faveur de la sécurité collective. C'est le rôle des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide des Nations unies, pour lesquelles notre contribution obligatoire s'établit à 384 millions d'euros. C'est également le cas de notre action au sein des organisations internationales, comme l'OTAN ou l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux fins de défense collective avec nos alliés ou de non-prolifération, telle que l'organise le traité de non-prolifération, le TNP. Nos contributions à ce titre s'élèvent à 372 millions d'euros.

Cette action doit être renforcée. Je pense bien sûr à la diplomatie économique offensive que le Gouvernement entend promouvoir. J'ai entendu les observations de M. Cadic sur ce point ; je compte bien

dispositifs innovants pour dégager des financements et assurer la promotion du tourisme. Les acteurs y sont prêts, et c'est dans cette perspective que nous avons confié à trois

Notre réseau culturel et nos établissements scolaires à l'étranger sont un instrument essentiel du rayonnement et de l'influence de la France dans le monde. Vous m'avez beaucoup interrogé sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

au travers de l'abondement du Fonds pour le développement de la vie associative. Sur ces 25 millions d'euros, 2 millions d'euros seront consacrés spécifiquement au financement des associations

à la fois des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger et des parlementaires représentant les Français de l'étranger, sur le modèle des commissions existant en matière d'aide sociale versée aux Français de l'étranger. J'espère que ces précisions sur le dispositif

Notre diplomatie est active à Bruxelles, mais aussi dans toutes les capitales européennes, pour expliquer et mettre en oeuvre les lignes d'action arrêtées par le Président de la République : agir pour l'Europe souveraine, pour l'Europe unie, pour l'Europe démocratique. Vous le savez, nos investissements en faveur de la construction européenne ne sont pas supportés par le budget de mon ministère, mais ils revêtent une importance majeure et connaîtront de nouveaux développements. La ligne action européenne de ce budget est

je l'ai déjà fait en commission, que je n'ai pas l'intention de céder des biens emblématiques de la présence et du rayonnement de la France dans le monde. Pour autant, une optimisation

La construction d'une chancellerie franco-allemande à Khartoum en est un exemple, de même que les coopérations avec le Service européen pour l'action extérieure à Tbilissi et à Quito.

sur le budget du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Le budget pour 2018 est sécurisé. Le ministère a procédé en 2017 à des ordres d'achat à terme de 532 millions de dollars et de 34,6 millions de francs suisses, ce qui permet de couvrir

Nous avons également proposé la mise en place d'ordres d'achat à terme pluriannuels, qui permettraient de sécuriser de 50 % à 70 % des dépenses en devises prévisibles. Enfin, nous travaillons à l'actualisation de la convention qui nous lie à l'agence France Trésor ; la signature est prévue à la fin de cette année. C'est un travail que nous poursuivons avec beaucoup de détermination.

de temps hors de notre territoire pour constater que toutes les puissances renforcent aujourd'hui les moyens de leur politique étrangère. Dans la période instable que nous traversons, il ne peut y avoir de souveraineté sans un instrument diplomatique efficace,

Je dois en effet vous rappeler que nous ne pourrons pas poursuivre la séance au-delà de minuit trente, horaire de rigueur. En effet, la nuit n'a pas été ouverte par la conférence des présidents et la séance doit reprendre demain matin, dès neuf heures trente, pour des questions orales. Nous avons 19 amendements à examiner sur les crédits de la mission et sur l'article rattaché. Si nous ne l'avions pas achevée ce soir, leur discussion devrait être reportée à vendredi matin, avant l'examen des articles non rattachés.

Depuis de nombreuses années, notre diplomatie économique a développé les relations commerciales entre les États. Néanmoins, la diplomatie économique crée des systèmes de dépendance lorsque les pays concernés sont de niveaux de développement inégaux. C'est sur cette base particulièrement inégalitaire, voire postcoloniale, que se sont renforcées des pratiques inappropriées. Des entreprises accumuleraient un maximum de contrats publics à l'étranger,

En parallèle, il est nécessaire de renforcer notre diplomatie culturelle. La culture, heureusement, n'est toujours pas une marchandise. Elle est d'une grande influence dans le monde et nous devons la protéger.

nous sommes contraints de laisser de côté ces familles en difficulté. Cette amputation de près de 10 % du budget de l'AEFE contraint celle-ci à prévoir la suppression de plus de 500 postes d'enseignant titulaire détaché, soit 8 % des effectifs actuels. Le Président de la République et le Gouvernement nous annoncent que les budgets seront pérennisés en 2018 et en 2019. Cela signifie qu'il n'y aura pas rétablissement de tout ou partie des subventions Pour les établissements conventionnés, cela implique une hausse immédiate des frais d'écolage ou le déconventionnement. Si un nombre important d'établissements scolaires se déconventionnent, l'AEFE aura à faire face à des problèmes de trésorerie accrus et l'on peut tout imaginer quant à la survie de cette agence. De plus, cela représente une perte d'influence de la France, puisque près des deux tiers des élèves des établissements français de l'étranger sont des étrangers qui, du fait de leur éducation française, deviennent francophones et francophiles. De nombreux élus consulaires nous interpellent et nous font part de la vive inquiétude qui remonte du terrain. Ils protestent très justement contre cette mesure qui affecterait grandement le réseau d'enseignement français dans leurs circonscriptions. Cet amendement vise à rétablir la part des subventions qui a été supprimée. J'espère pouvoir compter sur le soutien de mes collègues sénateurs représentant les Français de l'Hexagone qui, pour leur part, bénéficieront d'une augmentation de 1,3 milliard d'euros du budget de l'enseignement en France. Les Français de l'étranger n'ont pas à subir un enseignement au rabais

Si un tel amendement était adopté, ce serait une excellente nouvelle pour cet opérateur. En effet, sa situation financière délicate le conduit à envisager la suppression de 180 postes en 2018 et une hausse de 6 % à 9 % de la participation forfaitaire complémentaire des établissements conventionnés,

à « notre capacité à rayonner, l'attractivité de la France, notre capacité à continuer à faire des affaires ou des échanges culturels ou scientifiques À plusieurs reprises, monsieur le ministre, vous avez également mis en avant l'excellence du réseau d'enseignement français à l'étranger, la qualité des enseignants et les résultats au baccalauréat

suppressions de postes d'enseignant titulaire, baisse des subventions, passage de 6 % à 9 % de la participation financière complémentaire des établissements en gestion directe ou conventionnés. Cette discordance entre le discours et les actes est très mal vécue par les Français de l'étranger, qui vous ont pourtant, par leur vote à l'élection présidentielle et aux législatives, largement accordé leur confiance.

Cette incompréhension est d'autant plus forte que le Gouvernement a fait de l'éducation la priorité de son action et que le budget de l'éducation nationale a augmenté de 1,3 milliard d'euros. Certes, comme nous le savons tous ici, l'AEFE, qui existe depuis maintenant près de trente ans, a besoin de se réformer. Le rapport que j'ai présenté en 2014 avec le député Philip Cordery présentait déjà plusieurs pistes.

Monsieur le ministre, afin que le réseau de l'enseignement français à l'étranger continue d'être un outil d'influence incontournable pour notre pays, capable de former des personnalités aujourd'hui reconnues comme comme Amin Maalouf, Leïla Slimani, Jodie Foster, Carlos Ghosn ou Édouard Philippe- cette liste est loin d'être exhaustive -, il est indispensable d'abonder le budget de l'AEFE. C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de soutenir ces amendements.

fois la bourse scolaire déduite, est trop élevé par rapport à leurs revenus. Il convient donc, monsieur le ministre, de changer le barème.

Monsieur Le Gleut,

Cela a marqué une prise de conscience de l'exécutif des conséquences désastreuses de cette suppression, qui peut, dans certains cas, menacer la survie même des écoles françaises à l'étranger, des associations françaises à l'étranger, des Alliances françaises, de tous ces fleurons du rayonnement français à l'étranger qui bénéficiaient de la réserve

pour les réseaux culturels et d'enseignement français à l'étranger, pour nos associations qui accomplissent un travail remarquable et permettent que la voix de la France soit entendue dans le monde. Tel est l'objet de cet amendement, qui a été défendu à l'Assemblée nationale par notre collègue député Meyer Habib. L'amendement

Le réseau d'enseignement français à l'étranger, le réseau culturel des Alliances françaises, les différentes associations qui oeuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ont besoin de subsides publics Chaque année, la dotation d'action parlementaire a permis à mes collègues et à moi-même d'apporter un appui financier à ces structures. Pour ma part, je soutenais financièrement une cinquantaine d'associations à l'étranger, ce qui, au demeurant,

Il n'est pas concevable que cette aide s'arrête. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, monsieur le ministre, de revenir sur la décision de supprimer la réserve parlementaire, sachant que le Président de la République s'est engagé, le 2 octobre dernier, devant l'Assemblée des Français de l'étranger, à pallier les effets de sa suppression. Je ne saurais mettre en doute la parole du Président de la République, ni celle du Premier ministre, ni la vôtre, que vous avez donnée à l'Assemblée nationale. Je souhaite simplement, au travers de cet amendement cosigné par Claudine Lepage,

Mon lien avec le réseau des Alliances françaises est très étroit. J'ai en effet été administratrice de l'Alliance française de Dublin. J'ai aussi eu l'occasion de me rendre à des assemblées générales régionales annuelles, par exemple en Afrique du Sud, où s'étaient réunies les Alliances françaises Cet opérateur est un formidable outil pour notre rayonnement culturel, puisqu'il permet d'enseigner le français et de véhiculer notre culture à l'étranger. Néanmoins, en raison d'un héritage financier délicat, qui vient d'être rappelé, la situation de la Fondation Alliance française est critique : elle se trouve aujourd'hui confrontée à un déficit de trésorerie de 1,5 million d'euros.

Cette crise a été engendrée par les lourds investissements réalisés par la fondation dans le cadre de son plan stratégique quinquennal, le plan Alliance 2020, ainsi que par la non-perception de recettes locatives du fait du litige l'opposant à l'Alliance française Paris Île-de-France. Le ministère des affaires étrangères suit avec beaucoup d'attention la situation financière de la Fondation Alliance française, partenaire primordial pour la mise en oeuvre de sa diplomatie d'influence.

Par ailleurs, en plus de la subvention annuelle versée par le ministère à la fondation- d'un montant de l'ordre de 1,3 million d'euros -, l'État a apporté une aide exceptionnelle de 200 000 euros, imputée sur le fonds de dotation aux fondations et associations. la persistance des difficultés, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères vient de donner son accord pour que, de surcroît, 150 000 euros de crédits initialement destinés aux délégations générales de l'Alliance française soient réaffectés au fonctionnement de la fondation. Cela permettra notamment de régler les salaires de décembre 2017. Je précise que le réseau ne sera que très peu affecté par cette mesure, compte tenu de l'état suffisant de sa trésorerie pour faire face aux activités de la fin de l'année. L'État a d'ores et déjà apporté une contribution substantielle pour aider la fondation à traverser cette période critique. les conclusions du rapport des trois inspections, qui permettront d'objectiver les besoins réels de la fondation. Par ailleurs, nous suivrons avec la plus grande attention les résultats de la négociation en cours entre celle-ci et son principal partenaire bancaire. En tout état de cause, dans un contexte de raréfaction des crédits publics, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a engagé la fondation à reporter toutes les dépenses non indispensables et souligné la nécessité de prévoir des économies structurelles.

Le 27 septembre dernier a eu lieu une grève massive des enseignants français à l'étranger. Ils estiment, dans une déclaration commune, que le réseau des établissements français à l'étranger est clairement en danger. Une refonte du système de l'AEFE conduirait au déconventionnement de nombreux établissements, à la multiplication de formules éducatives au rabais, à la remise en cause de la situation administrative des personnels détachés et à la précarisation de l'ensemble des personnels. En réponse à ce constat très objectif, le Gouvernement ne propose que des rustines. La suppression des postes ne devrait pas toucher d'enseignants en cours de contrat : encore heureux, monsieur le ministre ! La La participation financière des établissements à la vie du réseau reviendrait à son cours actuel en 2020, ce qui signifie trois années de déstabilisation du réseau. C'est dire l'effet dévastateur de cette politique. politique. Un rapport permettrait de connaître les intentions réelles du Gouvernement, ses véritables motivations, ainsi que les solutions qu'il préconise pour remédier à la situation.

leurs parents. Privés de cette possibilité, ces enfants seraient petit à petit exclus du système d'enseignement français et auraient ensuite les plus grandes difficultés à intégrer les universités françaises. Les liens qui les rattachent à la France se distendraient de plus en plus. C'est bien souvent après s'être assurés qu'un établissement français pourra accueillir leurs enfants

l'avis de la commission ? Le problème soulevé est réel, mais il n'a pas paru opportun à la commission des finances qu'un opérateur puisse calculer son plafond d'emploi de manière dérogatoire.

effet un véritable problème d'équité entre catégories d'établissements. Néanmoins, la solution proposée n'est pas apparue opérante à la commission, notamment en

des établissements à la suite de la régulation budgétaire, vous proposez, monsieur Leconte, de créer une charge supplémentaire pour une catégorie d'établissements. J'ai un peu de mal à saisir